L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2021

En première lecture, nous avions pris acte de la mise à jour des données macroéconomiques du Gouvernement, en particulier de la très forte dégradation de nos finances publiques, avec un déficit public à 9,4 points de PIB et un endettement à 117,2 %. Le rebond Le rebond d'activité reste, quant à lui, fragile et serait moins important que celui de nos principaux partenaires européens. J'ai également émis de fortes réserves sur les reports opérés par le Gouvernement entre 2020 et 2021, qui atteignent un niveau exceptionnel cette année vont, à mon sens, bien au-delà de l'autorisation parlementaire. Enfin, il apparaît clairement que l'augmentation des dépenses prévue dans le présent PLFR répond à un objectif de précaution et de grande prudence. Pour autant, dès la première lecture, le Sénat a adopté, en responsabilité, les dispositions du collectif budgétaire tendant à accompagner la sortie de crise. Il en est ainsi de la prolongation, avec des adaptations, du fonds de solidarité ou encore la nouvelle aide au paiement des cotisations et contributions sociales. Le Sénat a également voté des mesures comme le renforcement du, qu'il appelait d'ailleurs de ses voeux depuis un an, ou encore la prolongation de l'octroi de la garantie de l'État au titre des prêts garantis par l'État, les PGE, et la reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, la PEPA. Le Sénat s'est montré constructif et raisonnable dans ses propositions de modification. J'en veux pour preuve les faibles évolutions de l'article d'équilibre à la suite de nos travaux. C'est ainsi que, outre des améliorations techniques et de sécurisation juridique, de nombreux apports du Sénat ont été conservés dans le texte adopté par la CMP, parfois à la faveur de compromis. Ce résultat est le fruit d'échanges fructueux avec nos collègues députés, en particulier avec le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, que je remercie de son écoute et qui a permis de rapprocher nos attentes. Ainsi, si j'ose dire, je suis globalement satisfait qu'un certain nombre de mesures aient pu rester dans le texte. Je ne les citerai bien sûr pas toutes- je vous renvoie au texte publié pour l'exhaustivité -, mais certaines méritent à mon sens d'être soulignées en ce qu'elles illustrent les objectifs que nous nous étions fixés pour l'examen de ce texte. Nous avons obtenu que la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, la PEPA, puisse être portée à 2 000 euros être exonérée d'imposition sur le revenu et de cotisations sociales, sans condition, pour toutes les entreprises de moins de cinquante salariés, et ce jusqu'au 31 mars 2022.

Dans le même esprit, et pour assurer l'équité fiscale, la commission mixte paritaire a maintenu l'exonération d'imposition sur le revenu votée par le Sénat pour la majoration exceptionnelle des indemnités de garde des internes perçues au cours de la première vague de l'épidémie. Nous avons également conservé plusieurs mesures permettant de soutenir les entreprises qui en ont encore besoin. Ainsi en est-il de l'exonération d'imposition de l'aide à la reprise des fonds de commerce perçue par les entrepreneurs ayant repris une activité au cours de l'année 2020, à l'instar de ce qui est prévu pour les bénéficiaires du fonds de solidarité, ou encore de la prolongation jusqu'à la fin de l'année 2022 du relèvement temporaire à 25 du taux de la réduction d'impôt applicable aux investissements dans les foncières solidaires chargées d'un service économique d'intérêt général, par parallélisme avec ce qui avait été voté à l'Assemblée nationale pour les souscriptions au capital des PME. En outre, la suppression du tarif réduit de TICPE applicable au gazole non routier a été reportée au 1janvier 2023. Nous sommes ainsi revenus à ce qui avait été annoncé par le Gouvernement. Les secteurs concernés

Nous sommes aussi venus en soutien aux collectivités territoriales en votant, par exemple, l'extension aux régies départementales du dispositif de compensation des pertes d'épargne brute, ainsi que la reconduction pour 2021 des « filets de sécurité applicables à certaines ressources spécifiques aux collectivités territoriales d'outre-mer et à la collectivité de Corse. Nous avons maintenu l'abattement dérogatoire à la taxe locale sur la publicité extérieure, issu d'un amendement de Nathalie Delattre,

Par ailleurs, la commission mixte paritaire a retenu deux ouvertures de crédits du Sénat au titre du plan de relance et directement destinées à l'action territoriale. D'une part, 10 millions d'euros supplémentaires sont consacrés à la forêt, afin que les travaux préalables à la reforestation entrent dans le champ des actions subventionnées, compte tenu des coûts parfois très élevés induits par de telles opérations à vocation environnementale.

D'autre part, et comme le demandait le président Claude Raynal, 50 millions d'euros supplémentaires sont affectés aux opérations d'investissement des AOM, les autorités organisatrices de la mobilité. Enfin, la commission mixte paritaire a adopté deux mesures tendant à mieux contrôler l'usage des crédits ouverts dans le cadre du PLFR. Cela concerne les crédits ouverts pour abonder le compte d'affection spéciale « Participations financières de l'État ainsi que l'enveloppe exceptionnellement élevée de la dotation pour « dépenses accidentelles et imprévisibles », à hauteur de 1,5 milliard d'euros. Je profite de ces quelques instants pour vous rappeler, madame la secrétaire d'État, qu'une solution doit être trouvée pour aider les entreprises créées en 2020 et qui, faute de chiffre d'affaires déclaré, n'ont pu obtenir aucun soutien de l'État. De même, le décret d'application doit permettre de faire entrer dans le dispositif de l'article 10 les quelques régies nouvellement créées et qui n'ont pas de perte d'épargne brute à déclarer. C'est parfois le cas dans certaines intercommunalités. Bien sûr, mes chers collègues, des regrets subsistent pour n'avoir pas su convaincre du bien-fondé de certaines mesures, comme celles qui visent à soutenir l'investissement dans la transition énergétique des entreprises. En tout état de cause, le PLFR se trouve indubitablement enrichi à la suite de son examen par le Parlement, notamment par le Sénat. Une fois l'activité repartie, il faudra mettre fin à l'économie « sous perfusion » des aides de l'État. Dès à présent, il faut aussi regarder vers l'avenir et déterminer une stratégie de redressement de nos finances publiques. notre inquiétude grandit, mais j'aurai l'occasion d'en reparler dès jeudi dans cet hémicycle, à l'occasion de l'examen du projet de loi de règlement pour 2020 et, surtout, du débat d'orientation des finances publiques,

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est un vrai plaisir pour moi de m'exprimer devant vous, en lieu et place de mon collègue Olivier Dussopt, qui, pour des raisons strictement budgétaires, a dû se rendre à Matignon. Il s'excuse platement auprès de vous de son absence.

rectificative pour 2021. Je tiens à le souligner, le texte dont nous débattons aujourd'hui illustre l'attachement du Gouvernement et des parlementaires à accompagner l'ensemble des acteurs économiques jusqu'à la fin de la crise sanitaire et à soutenir

ce collectif budgétaire est de financer l'accompagnement et le soutien à l'économie dans la sortie des mesures d'urgence déployées depuis le début de la crise liée au covid-19. C'est la raison nous vous avons proposé d'ouvrir 15,5 milliards d'euros de crédits pour prolonger les dispositifs de soutien bien connus des Français. Pour ce faire, nous vous avons proposé de provisionner 4 milliards d'euros pour les exonérations de cotisations et les aides au paiement 3,4 milliards d'euros pour le fonds de solidarité ; 6,4 milliards d'euros pour l'activité partielle, notamment l'activité partielle de longue durée. En outre, afin de prolonger l'aide aux secteurs privés d'activité, la mission « Plan d'urgence » est abondée de 150 millions d'euros supplémentaires pour financer les mesures au bénéfice du secteur de la culture. Le PLFR proposait initialement une série de nouvelles mesures pour mieux accompagner les Français et les entreprises jusqu'à ce que le chapitre de la crise soit enfin définitivement clos. Vous les avez enrichies tout au long de la navette parlementaire, ainsi qu'en commission mixte paritaire. Avec votre soutien,

renouvelons la prime « Macron » pour le pouvoir d'achat, qui permet aux entreprises de verser une prime exonérée d'impôts et de cotisations sociales pouvant s'élever jusqu'à 1 000 euros. Ce plafond sera porté à 2 000 euros pour toutes les entreprises de moins de cinquante salariés, grâce à l'assouplissement voté par le ainsi que pour les autres entreprises qui auront mis en oeuvre un accord d'intéressement ou qui s'engageront formellement dans des actions de revalorisation des travailleurs de la deuxième ligne. La prime pourra être versée jusqu'à début 2022 et la défiscalisation sera rétroactive, pour faire en sorte que les primes versées à partir du mois de juin puissent entrer dans le dispositif. Cette mesure doit rester exceptionnelle pour être pleinement efficace. Nous renforçons aussi

totalement déplafonnés. En outre, le texte issu de la CMP fixe au 1 janvier 2023 l'entrée en vigueur de la hausse des tarifs de taxe intérieure de consommation sur le gazole non routier. Cette hausse, qui devait initialement intervenir le 1 juillet dernier, aurait mis les entreprises concernées en grande difficulté, alors que les conséquences de la crise sanitaire se font toujours sentir. Enfin, s'agissant des aides et des dispositifs fiscaux relatifs aux entreprises, le texte de la CMP intègre la prorogation du taux majoré de la réduction d'impôt sur le revenu

Il en va de même pour le volet de ce dispositif dédié aux entreprises solidaires d'utilité sociale, les ESUS, dont nous connaissons tous, moi tout particulièrement, le rôle essentiel J'en profite pour les saluer. La deuxième responsabilité de ce collectif budgétaire est de prolonger le soutien aux collectivités territoriales, avec de nouvelles mesures attendues et ambitieuses. Nous vous avons donc proposé d'ouvrir 203 millions d'euros de crédits pour compenser les pertes financières enregistrées par des équipements gérés en régie qui n'ont pas pu être aidés jusqu'à présent. Les députés ont étendu le dispositif aux équipements gérés de manière déléguée, et vous l'avez vous-même étendu aux régies départementales du même type. Cette mesure parachève le dispositif massif de soutien aux collectivités territoriales depuis le début de la crise. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a inclus en première lecture dans le « filet de sécurité » des recettes du bloc communal pour cette année une compensation de la baisse des recettes du versement mobilité pour Île-de-France Mobilités. Cela était déjà prévu pour les autres autorités organisatrices de la mobilité.

ce PLFR renforce les facultés données aux élus locaux d'accompagner les acteurs économiques de leur territoire en prolongeant la possibilité offerte en 2020 au bloc communal de mettre en place à titre dérogatoire un abattement à la taxe locale sur la publicité extérieure. extérieure. La troisième ambition de ce PLFR est de faciliter le déploiement du plan de relance dans l'économie pour créer les conditions de la reprise au plus vite. Pour favoriser un engagement rapide du plan de relance, nous souhaitons ainsi réallouer 600 millions d'euros pour financer les dispositifs « Industrie du futur qui ont connu un fort succès, et grâce auxquels 8 500 projets au moins auront été financés. Un important volet de mesures nouvelles portées par ce PLFR concrétise en outre les priorités identifiées par le Gouvernement. Je ne reviens pas sur le détail des crédits ouverts

que le « quoi qu'il en coûte » nous permet certes de renouer avec l'activité rapidement, mais, vous le savez, il n'est pas sans conséquence. Le « quoi qu'il en coûte » n'aurait pu être mené à tout prix. Nous tenons toujours à restaurer l'équilibre qui a permis de répondre à la crise. Une fois la crise sanitaire passée, nous aurons besoin, faut-il le rappeler, surtout devant vous, d'un retour à la normale de nos dépenses publiques. Je ne pouvais éviter de le mentionner. La parole

je me réjouis que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord sur ce projet de loi de finances rectificative pour 2021. Néanmoins, le contenu de ce texte n'a rien de réjouissant. Il entérine en effet une situation des finances publiques des plus préoccupantes le déficit public s'est creusé de façon abyssale et le taux d'endettement s'est envolé. Ce n'est pas une surprise, simplement le résultat de la crise, dont nous continuons à payer le lourd tribut. Depuis le premier PLFR de crise, en mars 2020, la situation n'a cessé de se dégrader, et le rétablissement des finances publiques demeure une perspective encore très lointaine. À court terme, seule la croissance peut nous apporter quelques consolations, même si elle se mesure par rapport à une production nationale qui s'est effondrée en 2020. Néanmoins, elle est actuellement soutenue, et nous devons tout faire pour qu'elle le demeure. C'est le sens de ce PLFR. Au-delà de ces indicateurs, qui révèlent un tableau assez sombre, ce texte comporte de nombreuses mesures qui permettront de revenir progressivement vers une croissance durable.

dernière somme servira essentiellement aux travaux de renouvellement forestier, dont les coûts sont souvent très élevés. Ces crédits viendront renforcer ceux qui sont déjà prévus dans le plan de relance et combler des angles morts du dispositif actuel. Je tiens à saluer la mobilisation du rapporteur général sur ce sujet.

Je me réjouis également que le Sénat ait été entendu sur plusieurs propositions qui apportent des solutions concrètes à nos territoires. Cela vaut aussi pour les régies départementales, qui bénéficieront désormais du dispositif de compensation des pertes d'épargne brute. Enfin, je me félicite de l'accord trouvé sur la fiscalité du gazole non routier. Si notre groupe s'est rangé à la suppression programmée du tarif réduit de TICPE, nous considérons qu'une trajectoire plus progressive était absolument nécessaire dans un tel contexte de crise, où les entreprises ont besoin de stabilité réglementaire et fiscale. Au Sénat, nous avons été nombreux à relayer ces revendications, qui nous semblent légitimes. Il s'agit ici de trouver le juste point d'équilibre entre relance économique et transition écologique, dans la situation dégradée que nous connaissons.

sont versées parfois avec beaucoup de suspicion. Dernier exemple en date : Mme Vidal a annoncé la fin du repas à 1 euro dans les Crous, comme si les étudiantes et les étudiants n'avaient pas besoin de manger l'été ...

général Husson, mais les amendements de Joël Labbé, spécialiste du sujet, qui avait convaincu le Sénat de la nécessité de conditionner les aides du plan de relance au fait que les entreprises ne mettent en vente que du bois de chêne transformé au sein de l'Union européenne, et ce pour lutter contre l'exportation des grumes de chêne, ne sont plus

Nous avons fait toute une série de propositions afin de taxer davantage les plus riches, les multinationales. C'est pour nous une nécessité. Bercy a annoncé que l'impôt sur la fortune immobilière a rapporté 1,56 milliard d'euros en 2020, mais c'est toujours 2,5 milliards d'euros de moins que l'ISF

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, pour la première fois cette année, mais pour la cinquième fois depuis le début de la crise, nous nous retrouvons pour adopter définitivement un nouveau budget rectificatif, à l'issue d'une CMP conclusive qui nous aura permis d'enrichir le texte. Ce PLFR organise la sortie progressive des mesures d'urgence liées à la crise. Au total, ce sont près de 15,5 milliards d'euros de crédits destinés à prolonger les dispositifs de soutien 4 milliards d'euros pour le financement des exonérations de cotisations et des aides au paiement ; 3,4 milliards d'euros pour le fonds de solidarité et 6,4 milliards d'euros pour l'activité partielle, notamment de longue durée. Pour soutenir le secteur de la construction, nous avons reporté au 1 janvier 2023 la suppression du taux réduit de TICPE applicable au gazole non routier, conformément à l'engagement du Président de la République. La mesure a fait couler beaucoup d'encre. L'Assemblée nationale avait proposé de fixer au tout début de la prochaine législature cette suppression. je me félicite du rétablissement de ce report nécessaire, qui apporte un soutien bienvenu aux entreprises de nos territoires. Pour aider les entreprises toujours fortement touchées par la crise, y compris celles qui font l'objet d'une fermeture administrative, nous avons maintenu le dispositif fiscal de prise en compte des abandons de loyers et ouvert la faculté pour les communes de dégrever de taxe foncière les discothèques. Je me réjouis aussi de l'intégration, dans le filet de sécurité des ressources des collectivités territoriales pour 2021, des ressources spécifiques relatives à certaines collectivités d'outre-mer et à la collectivité de Corse, que le groupe RDPI a soutenue lors de l'examen en séance publique. Avec 50 millions d'euros de crédits supplémentaires ouverts en CMP pour compléter le financement des autorités organisatrices de la mobilité, un sujet notre président Claude Raynal s'était beaucoup mobilisé, nous renforçons avec efficacité le soutien massif apporté aux collectivités territoriales depuis le début de la crise. Le Gouvernement et les parlementaires accroissent également dans ce budget le soutien aux plus fragiles : 700 millions d'euros de crédits seront ainsi destinés au maintien du plan d'hébergement d'urgence hivernal pour toute la période estivale. C'est un effort considérable, qui permettra de laisser ouvertes 200 000 places d'hébergement jusqu'au mois d'avril 2022. Par ailleurs, 350 millions d'euros seront consacrés aux aides pour le secteur agricole après la période particulièrement difficile vécue en 2021. Nous voterons en outre avec ce PLFR une enveloppe de 100 millions d'euros pour financer le Pass'Sport, mais aussi 150 millions d'euros pour sécuriser le financement des bourses sur critères sociaux : autant de mesures en faveur de la jeunesse, qui aura payé un lourd tribut à cette crise. un mot de l'enveloppe de 1,5 milliard d'euros au titre de la dotation pour les dépenses accidentelles et imprévisibles, qui a été rétablie en CMP. Le groupe RDPI s'était fermement opposé à l'amendement qui visait à la réduire à 500 millions d'euros. L'ampleur de la crise justifie

au moins trois jours avant la publication de tout décret prévoyant le versement de plus de 100 millions d'euros sur un programme. Le pouvoir de contrôle du Parlement en est renforcé, et nous ne pouvons que nous en réjouir. À la lumière de ces différents ajouts, le groupe RDPI soutiendra par conséquent l'adoption de ce collectif

d'une forte reprise à l'automne. Notre espoir de revenir durablement à une situation normale réside essentiellement dans la vaccination à grande échelle, seule capable à ce jour de nous prémunir efficacement des effets les plus graves de cette maladie. Il semble que nous reviendrons sur ce sujet la semaine prochaine.

à renforcer les dispositifs de soutien à l'économie mis en place depuis 2020 : fonds de solidarité, chômage partiel, ou encore compensations au bénéfice de la sécurité sociale. Ces dispositifs ont permis, comme cela a été souligné en commission, d'absorber la plus grande partie du choc lié à la mise en sourdine de secteurs entiers d'activité. Les reports de crédits votés l'an dernier sont d'une ampleur exceptionnelle et ne correspondent pas à une situation budgétaire classique.

Le niveau de l'endettement public, quasiment à 120 % du PIB, reste préoccupant, même si la nouvelle dette contractée bénéficie de taux d'intérêt historiquement bas- mais pour combien de temps ? -et que le retour de l'inflation pourrait aussi limiter ses effets. dit, l'inflation pourrait précisément alimenter un rebond des taux. La charge de la dette augmente quand même de près de 1 milliard d'euros par rapport à la loi de finances initiale, début probable d'une augmentation qui va se poursuivre dans les prochaines années. En valeur absolue, le déficit serait de 220,1 milliards d'euros cette année, soit une dégradation de 46,8 milliards d'euros par rapport à la loi Il faudrait y ajouter le déficit de la sécurité sociale, qui devrait approcher 40 milliards d'euros pour la deuxième année consécutive. J'en viens maintenant aux mesures particulières.

La reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, exonérée de prélèvements sociaux, que les employeurs peuvent verser aux salariés permettra en particulier d'aider les salariés de deuxième ligne. Je salue surtout l'adoption définitive de l'amendement initialement déposé par mon groupe pour proroger en 2021 l'abattement à la taxe locale sur la publicité extérieure, de manière à permettre aux communes de soutenir les commerçants locaux. Enfin, les mesures de compensation de pertes de ressources offertes aux collectivités et à leurs établissements locaux devraient compléter utilement les aides qui avaient déjà été mises en place et qui comportaient, en vérité, quelques lacunes. En définitive, les membres du groupe du RDSE voteront pour l'adoption des conclusions de la

Et pour cause : comme chaque fois en de pareilles circonstances, nous nous réunissons au Sénat pour constater que vous avez négocié un texte au rabais. Il est à croire que nos travaux représentent finalement peu de choses

La majorité sénatoriale pourra également se réjouir du succès d'un amendement visant à reporter à 2023 la fin du tarif réduit de TICPE applicable au gazole non routier. Comme souvent, le Sénat s'arrime sur la position du Gouvernement. Il va même parfois plus loin que le groupe majoritaire La République En Marche de l'Assemblée nationale, qui demandait un moindre report de cette niche fiscale funeste pour l'environnement et extrêmement coûteuse pour les finances publiques. Alors que vous avez rejeté notre proposition d'accroissement des taxations sur les transactions immobilières supérieures à 1 million d'euros, je me dois de me borner à évoquer une proposition du groupe CRCE, adoptée par le Sénat, qui a finalement été répudiée dans le conclave de la

de taille intermédiaire et des grandes entreprises. Qu'une entreprise ne paye pas d'impôt sur les bénéfices lorsqu'elle est en déficit, c'est bien heureux, car elle n'en génère pas, mais qu'elle profite d'une créance fiscale au titre d'un exercice bénéficiaire du simple fait d'une mauvaise année, cela ne nous semble pas raisonnable. Ainsi, une entreprise structurellement bénéficiaire qui décide de racheter un concurrent pourrait se retrouver en situation de déficit et se faire rembourser l'impôt déjà versé. À nos yeux, c'est tout bonnement scandaleux ! Vous

cela reviendrait à permettre à un ménage de reporter ses créances causées par des dons d'argent aux membres de sa famille ou par des investissements dans sa voiture sur les années où il s'acquittait de l'impôt sur le revenu. Il en serait quitte avec de l'argent du fisc Nous n'avons pas vu l'opinion publique se mobiliser pour une telle demande, si ce n'est peut-être la majorité sénatoriale, qui s'enorgueillit de l'avoir proposée avant le Gouvernement. Il faut lire, le 28 mai dernier, pour comprendre vos intentions. Tout est dit dans le titre : « Report de déficits : un coup de pouce fiscal très attendu par les entreprises ». Voici la première phrase de l'article : « Un gouvernement au chevet des entreprises. la majorité présidentielle tout comme la majorité sénatoriale se fondent sur une croyance ainsi résumée dans le rapport de l'Assemblée nationale : « [ ...], si l'État renonce, à travers cet article, à des recettes fiscales contemporaines, il devrait recevoir, à l'avenir, des recettes fiscales d'entreprises qui seront restées à flot et renoueront avec les bénéfices. » Mais cela revient à nier la réalité ! Si les entreprises renouent avec les bénéfices, elles pourront, en cas de déficit, reporter en avant, sans limite dans le temps. Voilà ce qui risque de se produire : report en arrière, report en avant Voilà que vous sonnez- temporairement, nous dites-vous -la fin de l'impôt sur les sociétés. Mais vous trouverez bien une raison pour prolonger ce mécanisme d'allégement fiscal. Nous aurons peut-être droit un jour, mes chers collègues, au éternel ! La parole

Le groupe Union Centriste s'en réjouit. Depuis l'adoption conforme du premier budget rectificatif de mars 2020, au début de la crise sanitaire, c'est la quatrième fois consécutive que nous parvenons à une commission mixte paritaire conclusive sur un collectif budgétaire. Je pense que ce sens du dialogue et du compromis traduit tout simplement l'esprit de responsabilité des deux assemblées et du Gouvernement, ainsi que le respect des points de vue des uns et des autres, lorsqu'il s'agit de faire face à une crise sanitaire, économique et sociale de l'ampleur de celle que nous avons traversée. Il confirme aussi la capacité de dialogue des deux rapporteurs généraux- je tiens à le souligner. Désormais, chacun de nous espère évidemment que ce projet de loi de finances rectificative sera bien celui de la sortie de la pandémie, une sortie de crise marquée par la nécessité de poursuivre le soutien apporté par l'État, depuis près d'un an et demi, à nos concitoyens, à nos entreprises, mais aussi à nos collectivités locales. Sur ce dernier point, nous nous réjouissons vraiment de la compensation des pertes de recettes tarifaires au bénéfice de certaines communes fragilisées par la gestion de leurs services en régie. Le mécanisme retenu constitue une avancée importante, qui fait suite à l'engagement constant du Sénat sur ce sujet, ainsi qu'à l'engagement de M. le ministre Olivier Dussopt, que je tiens à remercier. D'autres motifs de satisfaction nous animent ; ils sont nombreux, à la hauteur des apports du Sénat conservés dans le texte final. Je veux rappeler une disposition en faveur des collectivités, que nous avons soutenue, sur l'initiative de notre collègue Sylvie Vermeillet : la réintégration dans l'assiette des opérations éligibles au FCTVA des dépenses engagées pour la réalisation, la modification ou la révision des documents d'urbanisme, ainsi que pour la numérisation du cadastre. C'est une disposition importante, en particulier pour les territoires ruraux,

Nous saluons aussi la prorogation jusqu'à la fin de 2022 du relèvement temporaire à 25 % du taux de la réduction d'impôt sur le revenu pour l'investissement dans les foncières solidaires chargées d'un service d'intérêt économique général. J'avais moi-même défendu un amendement en ce sens, et je suis heureux de la rédaction de compromis trouvée entre nos deux chambres. De la même façon, nous apprécions que la suppression du tarif réduit de TICPE applicable au gazole non routier soit bien reportée au 1 janvier 2023, comme votée au Sénat. Nous

Parmi les apports du Sénat et de sa commission des finances figure également la défiscalisation des rémunérations versées aux internes et étudiants en médecine au titre de leurs gardes. Cette mesure vient reconnaître leur engagement dans des conditions souvent difficiles, notamment au pic de la crise sanitaire. L'augmentation de 10 millions d'euros des crédits consacrés à la forêt par le plan de relance constitue un autre motif de satisfaction, particulièrement en effet compliquée pour la filière bois, en raison d'une convergence de facteurs qui la fragilise, alors même que son rôle est essentiel dans les réponses que nous devons apporter aux défis de notre temps. Bien sûr, quelques motifs de regrets demeurent. Nous avons bien entendu les explications concernant l'encadrement de l'exonération fiscale et sociale des aides du fonds de solidarité, qui se heurterait manifestement à un problème de sécurité juridique et au respect au respect du principe de confiance légitime. À n'en pas douter, d'autres propositions défendues par nos collègues du groupe Union Centriste auraient légitimement pu prospérer à l'issue de cette comme l'amendement de notre collègue Michel Canévet au sujet des dons familiaux, ou encore celui de Loïc Hervé visant à élargir le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante. Mais c'est la règle du compromis ; évidemment, nous l'acceptons. Malgré ces quelques regrets, notre regard demeure positif sur le travail effectué par les deux assemblées et sur l'accord obtenu. Aussi, la quasi-totalité du groupe Union Centriste approuvera les conclusions de cette commission

l'illusion d'avoir pris part à une discussion ! Pourtant, certaines mesures auraient largement mérité d'être retenues. J'y reviendrai tout à l'heure. Vous ne serez pas surpris non plus si je réaffirme que la politique menée par le Gouvernement depuis quatre ans ne nous convient pas. Alors que la fracture sociale s'amplifie, que la crise sanitaire creuse encore plus les inégalités et que les conséquences de cette crise affecteront durablement nos modes de vie les prochaines années, le Gouvernement maintient son cap. Parce que, pour nous, l'urgence sociale est une priorité, nous avions proposé un certain nombre de mesures visant à renforcer les services publics, qui sont le patrimoine commun de toutes les Françaises et de tous les Français. Ainsi, le plan d'urgence pour l'hôpital public proposé par le groupe socialiste tirait les conclusions de la crise sanitaire en lui redonnant les moyens nécessaires pour l'accueil et le suivi des patients, mais aussi en garantissant de meilleures conditions de travail pour nos soignants. Résolument tournés vers l'avenir, et pour laisser entrevoir de l'espoir à notre jeunesse, nous souhaitions aussi nous faire entendre sur la nécessité d'étendre le RSA aux jeunes Symbole de la précarité de notre jeunesse, les files d'attente d'étudiants pour l'aide alimentaire doivent nous interpeller et nous encourager à agir vite. Accompagner la jeunesse, c'est aussi donner les moyens nécessaires à l'éducation nationale. Après les annonces du ministre Blanquer, nous avons tenté d'encourager le Gouvernement à agir sans attendre pour engager la revalorisation du personnel enseignant, là encore en vain Nous avons aussi pu regretter l'absence de tout changement de doctrine fiscale, alors même que la crise a considérablement enrichi les plus riches de nos concitoyens et que certains grands groupes ont enregistré des profits record. À aucun moment, il n'a été envisagé de les mettre davantage à contribution ; ainsi, pas de rétablissement de l'ISF ni de hausse de la taxe sur les géants du numérique. Même l'OCDE nous invite pourtant à réfléchir à une fiscalité du patrimoine plus redistributive. Plutôt que de prendre ces sujets à bras-le-corps, le Gouvernement et la majorité sénatoriale ont préféré se réfugier derrière la hasardeuse théorie du ruissellement, alors que l'argent- il faut bien le constater -n'a jamais ruisselé. Ne pas envisager de recettes supplémentaires alors que le déficit se creuse et que la dette augmente est difficilement compréhensible, lorsque ne sont envisagées pour les réduire que la diminution de la dépense publique et la mise en oeuvre de réformes telles que celle des retraites. Nous savons bien toutes et tous ici à qui ces réformes porteront préjudice et à qui elles profiteront. Nous pensons qu'une autre voie est envisageable. Puisque la pédagogie est affaire de répétition, l'occasion nous sera donnée, lors de la discussion du prochain projet de loi de finances, de nous montrer particulièrement pédagogues. Mais nous sommes là sur des divergences de fond et même des divergences de convictions. On peut comprendre qu'il y ait des désaccords ; sinon, nous siégerions tous sur les mêmes travées. Pour autant, s'il y a bien un sujet sur lequel un consensus très large s'est dégagé au sein de notre assemblée, c'est pour soutenir une cause érigée au rang de priorité nationale : la lutte contre les violences faites aux femmes. Lors de nos discussions, notre assemblée, dans sa très grande majorité, a voté les amendements du groupe socialiste notamment celui qui, pour 2 millions d'euros seulement, visait à renforcer les crédits du 3919 et à conforter les moyens financiers des acteurs de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Qu'on ne nous fasse pas croire que la raison de ce blocage est simplement budgétaire ! La commission mixte paritaire n'a pas cru bon de devoir les retenir, souscrivant ainsi à la règle du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale refusant tous les amendements de crédits. Cependant, mes chers collègues, je suis convaincue que toute règle peut ou doit avoir des exceptions. En l'espèce, le nombre de femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint ne cesse d'augmenter. Il est de notre responsabilité collective de tout mettre en oeuvre pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Il y a, mes chers collègues, des occasions manquées qui sont lourdes de conséquences.

le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, modifié par lettre rectificative, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

acte la prolongation du dispositif SRU. À cette occasion, il s'agit de rechercher un équilibre entre obligation et adaptation locale, entre souplesse et contrainte.

Gouvernement. La commission a modifié l'équilibre de l'article 16 en exonérant de prélèvement SRU les communes qui touchent la DSR, en introduisant de nouvelles dépenses déductibles- de mon point de vue, ces dernières ne sont pas directement liées à la construction de logements sociaux

avec la construction de logements sociaux. C'est le cas pour les coûts d'éviction résultant des acquisitions foncières, ajoutés par la commission. En revanche, il nous semble que ce n'est pas le cas des coûts engendrés par la réalisation d'équipements qui serait rendue nécessaire par la construction de ces nouveaux logements et l'augmentation de la population qui en résulte. Concrètement, l'application de cette mesure serait sans doute source d'interprétation. Les besoins en nouveaux services s'apprécient à l'échelle de toute une population, pas nécessairement au regard de la construction de logements sociaux. Le produit des sommes recouvrées dans le cadre du prélèvement SRU est, par ailleurs, utilisé pour financer des acquisitions foncières et immobilières pour d'autres programmes de logements sociaux. Par souci de cohérence, notre amendement vise à en rester à la déduction des sommes effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian,

Alors que nous avons assisté à une augmentation des violences sexistes et sexuelles pendant la crise, nous sommes convaincus qu'il faut distinguer ces deux champs, qui correspondent tous deux à des besoins totalement différents. En effet, l'hébergement des femmes victimes de violence, par exemple, ne peut être cantonné à la simple question du logement social ; il s'agit d'un accompagnement global. Plus largement, l'hébergement d'urgence a besoin de davantage de moyens, ce que demandent depuis des années les associations, notamment les mouvements de protection des femmes et des mouvements féministes. Nous n'allons pas en ce sens en ne reconnaissant pas ce champ du logement social comme un

nous relevions qu'en 2018 cette exonération avait représenté un coût pour les communes de 500,4 millions d'euros, qui n'a été compensé qu'à hauteur de 16,2 millions d'euros de la part de l'État,

cet amendement vise à intégrer dans l'utilisation de l'amende SRU la possibilité de financer des travaux et équipements liés à la résilience et

Nous avons voulu prendre en compte les demandes légitimes de communes rurales, de communes d'Île-de-France et, plus généralement, de maires à qui le Gouvernement demande de faire

communes ont subi des catastrophes naturelles particulièrement traumatisantes, lesquelles n'ont pas épargné les logements sociaux et leurs habitants. Nous devons, bien évidemment, mobiliser le maximum de moyens pour prévenir de tels événements. Je suis parfaitement consciente que cela n'avance pas au rythme souhaité

le remplacement de la recette de taxe d'habitation est une fraction de taxe foncière et comme les constructeurs de logements sociaux ne supportent aucune taxe foncière pendant les vingt-cinq premières années, les communes qui voient arriver en 2121

Nous devons donc poursuivre l'effort de mixité porté par cette loi. Nous entrons en effet dans une période de grande fragilité sociale. Nous regrettons que deux de nos amendements aient été déclarés irrecevables. En effet, nous considérons que la suppression de la date butoir de 2025 conduit, en réalité, au travers des baux glissants, à repousser toujours plus loin le respect des objectifs, notamment pour les communes les plus déficitaires. Ainsi, le présent article prévoit que, pour l'ensemble des collectivités qui sont à moins de 4 points de leurs objectifs, soit près de 70 % des communes soumises à la loi SRU, l'effort à produire est de 33 %. Pour celles qui sont situées entre 4 et 2 points, l'effort serait porté à 50 %. Ces objectifs nous semblant peu ambitieux, nous proposions de les rehausser. Par ailleurs nous proposions de faire évoluer l'aspect qualitatif des objectifs de rattrapage. Les communes soumises à obligation de production de logements sociaux doivent produire seulement 30 de logements financés en PLAI et peuvent produire jusqu'à 30 % de logements financés en PLS. Nous souhaitons porter ces obligations à 50 % de PLAI et à 10 % de PLS. On ne peut ignorer qu'un million

pour l'attribution des logements très sociaux. Il faut donc poursuivre la production de ce type de logements pour répondre à la demande sociale. Vous l'aurez compris, pour nous, la souplesse apportée par ce nouveau dispositif ne doit en aucune manière

Nous proposons de rétablir le texte initial et de prévoir que l'objectif fixé par le préfet aux communes n'ayant pas atteint le taux de logements indiqué dans la loi SRU ne puisse être inférieur à ce taux. Il est essentiel pour nous de permettre, à titre dérogatoire, l'établissement d'un contrat de mixité sociale pour deux périodes triennales au maximum.

plancher, conformément à la jurisprudence de la cour d'appel de Versailles du 20 juin 2019, laquelle s'est fondée sur un faisceau d'indicateurs afin d'apprécier les freins à la construction de logements sociaux susceptibles de justifier l'abaissement des objectifs,

Ce contrat n'a pas vocation à devenir la règle. Nous considérons qu'il doit conserver son caractère temporaire d'adaptation des objectifs triennaux de rattrapage aux particularités locales. Les obligations en matière de construction doivent à terme rester identiques sur l'ensemble du territoire. Aussi, notre amendement tend à revenir au texte initial et à prévoir que le contrat de mixité sociale est conclu pour une durée maximale couvrant deux périodes triennales consécutives.

nous considérons que l'exercice des libertés locales, en l'occurrence des souplesses apportées à la loi SRU pour tenir compte des particularismes locaux et des difficultés spécifiques, doit se faire dans un cadre permettant une application unifiée des critères définis par la loi.

M. Didier Marie. Cet amendement vise également à rétablir l'avis préalable de la commission nationale SRU en cas de conclusion d'un contrat de mixité sociale qui déroge à l'objectif légal de rattrapage de réalisation de logements sociaux.

ne remet pas en cause l'objectif général. Je l'ai dit : le nombre de logements sociaux à construire n'est pas diminué, mais le rythme de rattrapage des communes déficitaires volontaires participantes sera lui fortement différencié. Nous sommes bien dans un texte qui traite de différenciation. La mutualisation ne se fera

coopératif et constructif avec l'État en faveur du logement social plutôt que de renvoyer les communes qui auront fait des efforts à leurs difficultés

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 1501, qui vise à rétablir l'échéance de 2025 et à supprimer un certain nombre de dispositions introduites en commission, dont la mutualisation intercommunale.

l'avis du Gouvernement ? Je partage évidemment le souhait d'une production équilibrée, notamment dans des grandes villes comme Paris, Lyon et Marseille. Toutefois, la loi prévoit déjà que le programme local de l'habitat, qui est un document opposable, opère une répartition des objectifs de production par arrondissement. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement, car contraindre la répartition des objectifs de réalisation au titre du présent projet de loi présenterait des difficultés de mise en oeuvre au regard de la prise en compte des situations locales et, surtout, de l'impossibilité juridique d'imputer les conséquences de la non-atteinte des objectifs à cette échelle.

Ces contrats favorisent certes un meilleur étalement dans le temps des objectifs, mais ils ne modifient jamais les objectifs chiffrés, rigides, alors qu'il est flagrant, nous le savons,

veulent et doivent construire des logements sociaux, mais en tenant compte des réalités. Ces réalités ont été peu prises en compte dans la loi SRU.

dans le décret du 5 mai 2017, les obligations de l'article 55 de la loi SRU sont trop contraignantes pour les communes touristiques, qui sont elles-mêmes soumises à des réglementations très rigides. zones inconstructibles, à la loi Montagne ou aux zonages de protection réglementaire comme Natura 2000. Les maires des communes touristiques souhaitent donc que l'État reconnaisse les particularités propres à leurs

L'effort de rattrapage contraint les élus locaux à réserver la délivrance des permis de construire à la construction de logements sociaux. L'article 17 du projet de loi modifie les seuils applicables aux communes nouvellement concernées par ces obligations, en prenant en compte les difficultés objectives éprouvées par les élus locaux pour effectuer ce rattrapage. C'est pourquoi cet amendement vise à rendre plus progressif le rythme d'entrée dans le régime d'obligation concernant les seuils de logements sociaux, en ajoutant une période triennale d'étape avant l'atteinte de l'objectif final et en fixant un point de départ plus raisonnable. Il est également proposé de conserver la possibilité de recourir aux contrats de mixité sociale.

d'obligation en matière de logements sociaux. Il apparaît que de nombreuses communes franchissent temporairement le seuil de population qui déclenche l'entrée dans le régime obligatoire. cet amendement vise à retenir une période triennale pour le constat du dépassement de seuil, ce qui permet de vérifier qu'une commune est entrée de façon pérenne dans le régime obligatoire.

le texte issu des travaux de la commission prévoit la signature obligatoire du contrat de mixité sociale par tous les organismes de logement social présents dans le département, ainsi que par les établissements publics fonciers.

ainsi que les engagements pris par les collectivités pour atteindre ces objectifs. Parmi les engagements devant être déterminés par ces contrats figureraient ceux en matière d'attribution de logements locatifs aux publics prioritaires. Le présent amendement vise à supprimer cette référence dans un souci de simplification de l'action publique locale. Plusieurs documents définissent déjà

et les établissements publics fonciers signent également le contrat de mixité sociale.

territoire. Un copilotage de ces contrats par les présidents de conseil départemental volontaire, aux côtés du représentant de l'État, pourrait donc être prévu. En effet, les départements qui sont d'ores et déjà délégataires des aides à la pierre sont engagés depuis de nombreuses années en faveur d'une politique de l'habitat équilibrée et adaptée aux besoins de chacun des territoires qui les composent. Autoriser le copilotage des contrats par le président du conseil départemental et le préfet de département est de nature à permettre aux communes et aux EPCI concernés de bénéficier de l'expertise et de l'appui en ingénierie des départements. C'est également de nature à favoriser la conclusion de contrats sur un périmètre comprenant éventuellement plusieurs intercommunalités, lorsque cela s'avère pertinent au regard des besoins du territoire.

Mme Dominique Vérien. L'un des objectifs visés par la construction de logements sociaux dans les communes est de favoriser la mixité entre leurs habitants.

L'impératif de mixité géographique et sociale est donc malheureusement compromis dans ces quartiers, qui sont souvent condamnés à vivre en vase clos, en partie du fait de leur éloignement des centres-villes.

ailleurs, pour éviter le phénomène bien connu de concentration de logements sociaux dans un seul et même quartier, le présent amendement vise à garantir une répartition équitable des logements sociaux sur la totalité du territoire communal,

mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence, dans notre tribune d'honneur, d'une délégation du Gouvernement de la Côte d'Ivoire. composée de M. Emmanuel Esmel Essis, ministre auprès du Premier ministre, chargé de la promotion de l'investissement privé, et de M. Roger Félix Adom, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, avec Son Excellence M. Maurice Bandaman, ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Paris. La délégation est accompagnée par notre collègue André Reichardt, président du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest. En visite en France, ils ont participé au colloque économique organisé au Sénat en partenariat avec Business France sur la Côte d'Ivoire, en présence d'une centaine d'entreprises françaises présentes en Côte d'Ivoire ou intéressées par les opportunités du marché ivoirien. Notre relation bilatérale avec la Côte d'Ivoire s'est renforcée au cours des dernières années, ancrée dans l'histoire et le partage de la francophonie. La création récente d'un Sénat en Côte d'Ivoire nous a permis d'intensifier notre coopération interparlementaire, qui a pris corps dans le cadre d'un accord visant à accompagner le Parlement ivoirien dans la mise en place du bicamérisme. Mes chers collègues, en votre nom à tous, permettez-moi de souhaiter à nos amis ivoiriens la plus cordiale bienvenue au Sénat français. Nous reprenons

de non-automaticité et de proportionnalité des sanctions pour carence, et ce afin de respecter le principe de libre administration des collectivités territoriales figurant à l'article 72 de la Constitution.

prélever un certain nombre de sommes, parce qu'elles n'auraient pas atteint leurs objectifs. Je rappelle que la commission a par ailleurs supprimé toutes les sanctions qui ont été jugées inutiles et contre-productives. Quel est l'avis du Gouvernement ? Le

réduction des sanctions possibles, alors même que le rapport de la commission nationale SRU, rendu en janvier 2021, conclut que la pérennisation des objectifs de la loi SRU doit s'accompagner d'une « fermeté accrue »

Nous considérons que ces outils sont utiles et doivent permettre au représentant de l'État de prendre des mesures concrètes, à charge pour lui de s'en saisir pour négocier avec la commune.

auprès du représentant de l'État dans le département à poursuivre cet effort sur les deux années suivantes bénéficient d'une réduction de la pénalité appliquée au titre de la loi SRU et échappent aux sanctions en matière de gestion des permis de construire et des attributions de logements sociaux.

La demande accrue de résidences secondaires augmentant le prix du foncier et des logements disponibles à la vente, la population permanente locale ne se trouve plus en mesure d'acquérir une résidence principale à un prix raisonnable, en adéquation avec le pouvoir d'achat local. Dans ces zones tendues de montagne, la collectivité locale ayant la compétence en matière d'urbanisme pourrait mettre en place une zone de protection de l'habitat permanent dans le PLU. Cette zone protégée viserait à réserver, en priorité, le foncier disponible ainsi que les constructions déjà existantes à l'accession principale, afin d'y maintenir la population locale, garante d'une activité économique à l'année. La collectivité locale pourrait également instaurer une taxe annuelle liée à toute modification d'usage de la résidence principale. Tel est l'objet de cet amendement. Quel est l'avis de la commission des affaires